La séance est reprise. J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique a été publiée. Cette candidature sera ratifiée si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement.

Dans la discussion générale, la parole est à M. Emmanuel Capus, auteur de la proposition de loi. Monsieur

avoir échangé avec la commission des lois, notamment son rapporteur François Bonhomme, dont je salue la qualité du travail, il nous est apparu

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi d'Emmanuel Capus a été déposée en quelque sorte en réaction aux élections européennes de mai dernier. Elle vise à mieux accompagner les maires dans la gestion de la propagande électorale, alors que beaucoup ont manqué de panneaux pour apposer les affiches des trente-quatre listes- pas L'obligation d'installer des panneaux électoraux remonte à une loi bien lointaine, datant de 1914. Il s'agissait déjà, à l'époque, de garantir une certaine équité entre les candidats. Le rapporteur

Ces panneaux métalliques sont aujourd'hui installés pour l'ensemble des scrutins, à l'exception des élections sénatoriales. Comme pour la tenue des bureaux de vote, les communes agissent au nom de l'État, qui leur verse en contrepartie une dotation pour frais d'assemblée électorale. Tous les candidats bénéficient d'une surface identique pour apposer leurs affiches. L'État rembourse les dépenses des candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix, généralement fixé à 5 % des suffrages exprimés. comme chacun a pu le constater, beaucoup de communes ont manqué de panneaux électoraux lors des dernières élections européennes. De nombreux articles de presse ont évoqué une « pénurie de panneaux », un « casse-tête logistique » ou encore des maires contraints de « bricoler » pour sortir de l'impasse. Je rappelle que les maires ont eu moins de dix jours pour trouver des solutions, incluant deux week-ends et un jour férié. En l'absence de rallonge financière du Gouvernement, ils ont dû recourir au « système D » en scindant leurs panneaux en deux parties, en fabriquant leurs propres panneaux ou en délimitant de nouveaux emplacements sur les murs des bâtiments publics. Cette situation paraît d'autant plus absurde que nombre de panneaux sont restés inoccupés.

En pratique, certains candidats n'impriment qu'un nombre réduit d'affiches, notamment lorsqu'ils ne pensent pas atteindre le seuil de remboursement de leurs dépenses. D'autres rencontrent des difficultés matérielles pour « approvisionner » les panneaux, malgré l'aide des militants.

À mes yeux, le retour à la circonscription unique a encouragé la multiplication des listes de candidats et créé des difficultés matérielles, qui n'ont pas été suffisamment anticipées.

proposition de loi aborde le problème sous un angle différent, en cherchant à rationaliser l'utilisation des panneaux électoraux. La commission des lois y est favorable : l'intervention du législateur peut permettre, je l'espère, de mieux accompagner les maires et d'éviter ainsi de s'en remettre au « système D ». Elle a donc adopté la proposition de loi, tout en sécurisant son dispositif et en préservant la liberté d'expression des candidats, qui constitue, je le rappelle, un droit de valeur constitutionnelle. Elle a également différé l'entrée en vigueur des dispositions du texte, pour éviter toute interférence avec les prochaines élections municipales. Au titre du premier mécanisme proposé, les candidats devraient préciser, dans leur déclaration de candidature, s'ils souhaitent ou non utiliser leurs emplacements. Le « droit aux panneaux » ne serait pas remis en cause pour autant. Tous les candidats pourraient en bénéficier, à condition d'en faire la demande en amont de la campagne. L'objectif est simple : éviter d'installer des panneaux inutiles, que les candidats ne souhaitent pas utiliser. Par ailleurs, la commission a supprimé le dispositif de sanction, qui lui paraissait à la fois complexe à mettre en oeuvre pour les maires et disproportionné pour les candidats. Elle a privilégié un système de déclaration sur l'honneur, qui reposera sur la bonne foi des candidats. candidats. Nous avons également instauré un « droit au remords ». Chaque candidat pourra solliciter l'installation de panneaux électoraux jusqu'au vendredi précédant le scrutin.

S'agissant spécifiquement des élections européennes, nous avons ajusté le calendrier du scrutin pour que les communes disposent d'une semaine supplémentaire pour installer leurs panneaux. Initialement, le deuxième mécanisme prévu dans la proposition de loi prévoyait de réduire de moitié le nombre et la dimension des affiches lorsque les panneaux électoraux sont utilisés par plus de quinze candidats. Ce dispositif soulevait toutefois quelques difficultés opérationnelles : pour des raisons calendaires, la taille des affiches ne peut pas être modifiée à quelques jours du scrutin. Dans un souci de compromis, la commission a proposé un mécanisme plus souple, consacrant la possibilité pour le maire d'adapter les dimensions des panneaux électoraux en fonction des circonstances locales.

À l'inverse, la dématérialisation n'est pas de nature à améliorer la participation des citoyens les plus âgés ou vivant encore dans des zones blanches. Le Gouvernement semble d'ailleurs avoir renoncé à cette idée, après trois échecs consécutifs devant le Parlement. J'espère, madame la ministre, que vous pourrez nous confirmer cet élément. À la suite de mes auditions, je dois alerter le Sénat sur les conditions d'organisation des élections régionales et départementales de mars 2021. En effet, les professionnels du secteur, que j'ai reçus avec Alain Richard,

doutent fortement de leur capacité à mettre sous pli et envoyer en temps et en heure l'ensemble des documents de propagande. Leurs inquiétudes concernent surtout le second tour : pour ces deux scrutins, les candidatures seront déposées le mardi soir, les commissions de propagande devront se réunir le mercredi et les envois devront être réalisés, au plus tard, le jeudi ou le vendredi. Peu réaliste, ce calendrier représente un risque pour l'acheminement des professions de foi jusqu'aux citoyens.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, notre droit électoral est fait de règles répondant toutes à un même principe : l'égalité de traitement entre les candidats. C'est le sens que nous donnons aux dispositions sur les bulletins de vote, sur la propagande télévisée et, bien sûr, également sur l'affichage. le principe : tous les candidats à un scrutin doivent disposer d'un emplacement d'affichage à proximité de chaque bureau de vote pour pouvoir y coller leur affiche de campagne. Cette règle, et je préfère le dire d'entrée, je la crois saine. Elle est une garantie pour chaque candidat ou liste de pouvoir bénéficier d'un affichage égal. Elle est l'assurance d'échapper aux luttes de collage qui peuvent exister sur l'affichage public. Elle est la certitude, pour tous ceux qui le souhaitent, d'être vus au moins une fois par les électeurs. Par cette proposition de loi, monsieur le sénateur Capus, vous soulignez une difficulté à laquelle les communes peuvent être confrontées une difficulté que j'entends parfaitement, étant ancien maire d'une commune de 4 500 habitants ; une difficulté, enfin, qui a été mise au jour lors des élections européennes de mai dernier. Il s'agit du nombre important de listes ou de candidatures- elles étaient trente-quatre, comme cela a été rappelé, aux élections européennes. Je me tourne tout de même vers le rapporteur pour faire observer que la participation aux élections européennes a été très au-dessus de la moyenne habituelle, ... Cela étant dit, il est parfois difficile pour les maires, notamment dans les petites communes, de se conformer aux exigences du droit, soit par manque de panneaux d'affichage, soit par manque d'espace sur la voie publique, voire les deux.

qui leur appartiennent et que nous n'avons pas à commenter, ont préféré limiter leur affichage et laisser vierges de nombreux panneaux. Cette difficulté, donc, je la comprends. Je l'entends. Elle appelle néanmoins, et avant d'aborder précisément le texte,

face à l'exceptionnel et accompagner les maires dans toutes les situations. C'est la raison pour laquelle une subvention pour frais d'assemblée électorale est mise en place à chaque scrutin. Elle vise à compenser les frais supplémentaires que les communes supportent pour l'organisation d'une élection. élection. Pour en venir plus précisément au texte, ses dispositions manquent, je le crains, leur objectif et risquent d'être inopérantes ou inapplicables. de loi, telle qu'elle a été modifiée par la commission, ne prévoit plus aucune sanction pour les candidats qui choisiraient de ne pas apposer leurs affiches, ou alors de les apposer seulement devant certains bureaux de vote. Il est à craindre que cette mesure retire les effets utiles du texte et que, par mesure de précaution, toutes les listes candidates déclarent leur intention de mettre des affiches et avisent ensuite sur quoi faire réellement. J'ajoute que le texte, dans sa rédaction actuelle, risquerait de provoquer des problèmes logistiques nombreux et, parfois, insurmontables pour les maires.

l'article 1 offre la possibilité aux maires de réduire la dimension des panneaux d'affichage, lorsque le nombre de demandes d'emplacement est supérieur au nombre de panneaux disponibles localement. J'y suis favorable, mais cet objectif peut être atteint par voie de circulaire sans qu'il soit nécessaire de légiférer et, donc, de rigidifier notre droit. Je ne prendrai que l'exemple des dernières élections européennes, pour lesquelles les maires avaient été autorisés, par circulaire, à scinder en deux parties égales les panneaux d'affichage en cas de besoin. Enfin, je crains que le texte ne fasse peser des contraintes trop fortes, voire insurmontables sur certains candidats ou certaines listes. La rédaction retenue à l'alinéa 8 de l'article 1 laisse à penser que le maire serait en mesure d'imposer aux candidats la taille des emplacements et, par conséquent, de leurs affiches, en cas de de manque de panneaux dans une commune. Cela pourrait provoquer des ruptures d'égalité et des contraintes extrêmement difficiles à supporter pour les candidats ou les listes : imaginons que, dans une même circonscription, il y ait plusieurs jeux de tailles d'affiches à prévoir. Mesdames, messieurs les sénateurs, ce texte met le doigt, justement, sur une question pouvant préoccuper les maires lors de certains scrutins. Je crois toutefois que nous avons tout à gagner à garder une forme de souplesse dans notre droit et de capacité à nous adapter aux circonstances de chaque élection, plutôt que de risquer de graver dans la loi des mesures dont nous ne pouvons pas avec certitude garantir les effets. C'est pourquoi je ne pourrai pas défendre ce texte, sur lequel le Gouvernement émettra un avis défavorable. La parole

ont voulu, de manière concrète, corriger et rationaliser un dispositif d'affichage électoral devenu un vrai casse-tête pour les mairies à l'occasion des élections européennes. L'obligation de mise en place de trente-quatre panneaux d'affichage, dont moins de la moitié a finalement été utilisée par les listes

deux autres arguments, qui n'ont peut-être pas été tellement mis en avant dans les débats en commission. Le premier est le problème de l'occupation du domaine public, surtout lorsque les panneaux ne peuvent pas être plaqués contre un mur ou une clôture. Dans le cas des élections européennes, il fallait tout de même un linéaire disponible d'au moins

de gaspillage inutile en termes de matériaux et de temps passé par les services municipaux, telle qu'elle peut être perçue par nos concitoyens. Je voudrais aussi rappeler qu'à l'origine l'affiche électorale était destinée à afficher le programme des candidats, même si elle a ensuite évolué vers un concept plus promotionnel de slogans, comme en témoignent les affiches exposées au sous-sol du Sénat, à proximité de la salle Clemenceau. Aujourd'hui, l'affiche n'a plus aucun impact pédagogique. Elle vise essentiellement des objectifs de marketing électoral, c'est-à-dire d'identification, d'attractivité, avec un éventuel message qui, pour être percutant, doit être le plus court possible. Dans ces conditions, aussi bien la multiplication des panneaux que la réduction de la taille des affiches ne sauraient répondre à l'exigence de lisibilité, donc d'utilité, de l'affichage électoral. mes chers collègues, que seule l'introduction d'un filtre permettant de limiter les candidatures à un nombre raisonnable de listes constitue la bonne solution dans le cas des élections européennes. À la suite de cet argumentaire, il me semble un peu difficile d'approuver certaines dispositions de l'article 1 de ce texte. Certes, la déclaration d'une intention d'utiliser un panneau d'affichage est une bonne mesure.

Cela pourrait être équitable pour un scrutin communal, mais pas pour les autres élections, qui se déroulent sur une circonscription plus large, comprenant des communes susceptibles de prendre des dispositions différentes en matière de taille de panneaux, donc de

Je voudrais évoquer deux autres sujets qui ne figurent plus dans le texte. Le premier concerne le grammage du papier pour les bulletins de vote et les circulaires- c'était l'article 2 du texte d'origine. Ce grammage est bien de 70 grammes. La disposition est confirmée par le décret du 27 décembre 2019, mais aussi par l'arrêté interministériel du 24 janvier 2020 concernant les tarifs de remboursement des frais d'impression des documents électoraux pour les élections municipales.

me paraît quelque peu ambigu. En effet, cet article ne serait satisfait que par exception, car les bulletins de vote doivent bien être fabriqués en 70 grammes pour être acceptés par la commission de propagande, diffusés et éventuellement remboursés.

Cela manque tout de même de cohérence. Il aurait donc été bien préférable de conserver l'ancienne disposition, permettant l'utilisation de papier de grammage compris entre 60 et 80 grammes, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est l'autoédition des bulletins de vote. dans ce cas-là, que la condition est satisfaite. La deuxième raison, c'est la sécurité d'approvisionnement des imprimeurs sur un papier qui n'est pas le plus utilisé- le 70 grammes donc avec des risques d'augmentation du prix du papier, voire de rupture de stock, le papier le plus générique demeurant l'80 grammes.

déclaration d'intérêts. Madame la ministre, c'est donc à vous que je m'adresse pour corriger l'arrêté du 24 janvier 2020 ou diffuser une circulaire recommandant une tolérance jusqu'à 80 grammes, afin de donner un peu de souplesse aux fournisseurs d'imprimés électoraux.

Sous le même titre, on pourrait peut-être à l'avenir effectuer un balayage plus complet, que ce soit sur le plan législatif ou réglementaire, pour moderniser un dispositif ayant accumulé au fil du temps imprécisions et incohérences, certaines étant bien récentes, comme celle que je viens d'évoquer sur le grammage du papier.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le débat de cet après-midi a un parfum de terroir. ! Nous évoquons des difficultés en milieu villageois, la réponse de bon sens de nos chers élus locaux ... Très bien ! Vous voyez le climat : c'est vivifiant

je voudrais aller plus loin, stimulé par le fait que François Bonhomme a souhaité rouvrir une querelle qui nous avait opposés durant le débat sur la réforme du mode de scrutin des élections alors parmi les plus ardents défenseurs du maintien du système par circonscriptions régionales. Ce débat a eu une particularité,

je n'avais pas eu le « cran », si j'ose dire, de présenter un amendement visant à instaurer, comme l'ont fait pratiquement tous nos voisins européens, un système de filtrage. En effet, si l'on regarde les autres élections, on n'a jamais trente candidatures. Quelle que soit la nature de l'élection, il y a toujours un facteur modérateur le nombre de candidats à trouver pour les élections municipales, la faible chance d'accéder au tour décisif pour les élections départementales, etc. Je ne multiplie pas les exemples,

pour accéder à ce financement modère tout de même le nombre de candidatures, quoique, en milieu urbain, notamment quand la circonscription est importante et apporte plus de voix, on atteigne parfois les dix-huit ou vingt candidats.

Donc, même si quelques dispositions organiques obligeraient à repasser directement devant le législateur- mais celui-ci peut être de bonne foi et ne pas détourner un débat de codification -, je pense qu'il faudra le faire. Je conclus en rappelant ce vers de Victor Hugo, que je ne sais plus situer

Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, je vous avoue que je suis à la peine, ... Déjà ! ... parce que, d'un côté, cette proposition de loi part d'une bonne intention : qui ne voudrait pas faciliter la vie des maires

sur ce problème à partir d'un cas particulier et, donc, tirer des leçons générales de ce cas particulier Faut-il complexifier encore un peu plus l'arsenal de régulation du droit électoral ?

On risque ainsi une multitude de contentieux et de difficultés avec les commissions de propagande, qui ne sont pas toujours cohérentes entre elles. Surtout, on risque on risque de limiter une nouvelle fois l'information non médiatisée, celle qui ne passe pas par les filtres médiatiques de l'élection, dont tout le monde s'accordera pour dire qu'elle est tout à fait essentielle.

où l'affichage militant est relativement important par rapport à l'utilisation de prestataires de services,

en essayant de régler des problèmes qui se posent lors des élections européennes, on risque, sans le vouloir, d'en créer de nouveaux dans d'autres situations.

le maire a dû faire installer pas moins de 102 panneaux électoraux, dont la moitié est restée sans affiche, ce qui a valu au maire les foudres de sa population, qui ne comprenait pas qu'on investisse dans des panneaux inutiles. Les maires ont eu le plus grand mal à se fournir en panneaux électoraux, et beaucoup d'entre eux ont dû organiser des sortes d'ateliers de bricolage, chez eux parfois, pour trouver des solutions de fortune.

Elle a le mérite d'épargner aux maires un certain nombre de migraines et l'installation inutile et coûteuse de panneaux électoraux. Je suis assez favorable à la proposition de ne fournir un panneau qu'aux seuls candidats qui en font la demande. Je comprends la réserve

la dimension des panneaux électoraux, je partage la volonté de souplesse et les conditions qui ont été prévues. Je salue aussi l'initiative du rapporteur sur le calendrier des élections européennes : dix jours ne suffisent pas lorsqu'il y a autant de candidats.

l'affichage de la propagande électorale et les bulletins de vote imprimés à domicile. Le second volet a été retiré du texte, puisqu'il est satisfait par un décret de 2019. Le texte, Le texte, tel qu'il nous est proposé à la suite de son examen en commission, s'attache donc à la seule question de l'affichage. Comme cela a été largement souligné, les maires ont l'obligation d'installer des emplacements dédiés à ces affiches,

l'information égale de chacun, la défense de toutes les opinions et l'égalité, qui est un principe constitutionnel, entre les candidats. La proposition initiale

le candidat. Or sécuriser l'organisateur et éviter une insécurité juridique est tout de même l'objectif du texte. En ce sens, la suppression du régime de sanction proposée par le rapporteur et adoptée en commission nous paraît plutôt une bonne chose. Le régime de déclaration permet à tous de bénéficier de panneaux, à condition d'en faire la demande. L'égalité entre les candidats est donc garantie, et ce d'autant plus que le texte issu de la commission instaure un droit au remords qui permet, jusqu'au dernier moment, d'utiliser ce panneau. Au-delà de la question des panneaux d'affichage se pose celle de la taille des affiches.

avec autorisation d'apposer les affiches, alors que la clôture du dépôt de candidature est le 27 février, à dix-huit heures, soit trois jours avant, ce qui pose de manière évidente des problèmes de délais. La proposition par le rapporteur, qui a été très créatif, comme les maires sur le terrain, et à laquelle nous souscrivons, est de mettre en place un système autorisant le maire à adapter les dimensions des panneaux si plus de quinze candidats se présentent et en respectant le principe d'égalité entre les candidats. Au final, c'est le maire qui a le droit d'adapter les modalités et pas le candidat qui est contraint. contraint. En termes de régime juridique, ce n'est pas plus mal. En l'état des modifications adoptées par la commission des lois, ce texte ne pose pas de problème juridique particulier. Il a le mérite de sécuriser le maire, ce qui était le but recherché. En ce sens, il peut être considéré comme utile, même s'il n'apporte pas grand-chose et que, selon les propos de Mme la ministre, il a peu de chance d'aboutir. Pour permettre aux maires de continuer à faire oeuvre de créativité, nous le voterons ! Très

voterons ! Très bien ! La parole est à M. Cyril Pellevat. Monsieur le rapporteur, François Bonhomme, je tiens tout d'abord à vous remercier et à vous féliciter pour le travail que vous avez fourni, ainsi que pour vos conclusions sur la proposition de loi relative à la simplification et à la modernisation de la propagande électorale, la ministre, mes chers collègues, ce texte vient tirer de nécessaires leçons des élections européennes de 2019 et a pour but d'accompagner au mieux les maires dans leurs obligations d'installation de panneaux électoraux et de gestion des bulletins de vote. proposition de loi est tout à fait profitable en ce qu'elle permet de pallier les problèmes qui apparaissent avec la multiplication des candidatures. En effet, cela a été rappelé, avec les trente-quatre listes présentées aux dernières élections européennes, de nombreuses communes ont été confrontées à un manque de panneaux, alors que la loi les oblige depuis 1914 à en installer pour chacune des listes. Afin de répondre à cette obligation, les maires ont dû trouver des solutions de dernière minute, sans augmentation de leur dotation et dans un laps de temps extrêmement court. Or, et ce malgré leurs efforts pour réunir un nombre suffisant de panneaux, qui ne peuvent être que salués, nous avons assisté à une désertion des panneaux par les candidats, nombre d'entre eux n'ayant pas les moyens d'imprimer des affiches s'ils n'atteignaient pas les 5 % de suffrages nécessaires au remboursement par l'État de leurs dépenses. Il n'est pas juste pour les communes que la loi leur impose de si lourdes charges sans augmenter leur dotation, alors même que les solutions qu'elles ont trouvées n'ont pas été utilisées. Il était donc nécessaire de trouver des solutions à ces dysfonctionnements. C'est l'objet de cette proposition de loi, dont je salue l'auteur, en rationalisant l'utilisation des panneaux électoraux ainsi qu'en assouplissant les règles de grammage des bulletins. bulletins. La proposition de loi impose désormais aux candidats de préciser dans leur déclaration de candidature s'ils souhaitent utiliser les panneaux électoraux, ce qui permet aux maires d'installer des panneaux non plus pour l'intégralité des candidats, mais uniquement pour ceux qui en font la demande.

Cet amendement prévoit également un « droit au remords » pour les candidats qui peuvent demander l'installation de panneaux jusqu'à deux jours avant le début de la campagne. Cela permettra plus de souplesse pour les candidats souhaitant modifier leur stratégie électorale en fonction des financements reçus ou de l'évolution des sondages. Cette proposition de loi prévoyait également de réduire de moitié le nombre et la taille des affiches des candidats dès lors que plus de quinze demandes d'utilisation des panneaux étaient déposées. Cependant, cette disposition serait difficile à mettre en oeuvre, de nombreux candidats étant contraints d'imprimer leurs affiches avant même de connaître le nombre total de candidats. C'est pourquoi un autre amendement a été adopté en commission, permettant plus de souplesse. Il consiste à donner la possibilité au maire d'adapter les dimensions des panneaux, à condition que le nombre de panneaux à installer soit supérieur à quinze, que la commune ne dispose pas de suffisamment de panneaux et que tous les candidats bénéficient de la même surface. de loi prévoyait d'assouplir les règles de grammage des bulletins de vote, afin de sécuriser l'impression par les électeurs de leur propre bulletin. Elle autorisait un bulletin pesant entre 60 et 80 grammes par mètre carré. Cela n'est toutefois pas nécessaire, car il existe déjà un décret en la matière. Cette possibilité pour les citoyens d'imprimer chez eux le bulletin de vote est bénéfique, car elle permet aux petits partis de ne pas utiliser leurs fonds pour réaliser eux-mêmes les impressions ; elle est également bénéfique d'un point de vue écologique. J'irais toutefois plus loin en matière de bulletins, car ces derniers sont imprimés par millions, alors que la quasi-totalité est détruite sans avoir servi. Il s'agit d'un véritable désastre écologique. J'ai donc en ce sens déposé une proposition de loi visant à instaurer un bulletin de vote unique, qui consiste à remplacer les bulletins de vote actuels par un bulletin unique sur lequel chaque candidat est inscrit. Les citoyens Les citoyens voteraient alors en cochant le candidat de leur choix sur ce bulletin unique, à l'image de ce qui se fait en Allemagne, en Belgique et aux États-Unis. L'impression et la distribution de ces bulletins seraient financées par l'État, mais leur coût, qui est estimé à 1,5 % du remboursement de la campagne par l'État, serait compensé par la baisse de l'enveloppe destinée au remboursement des frais de campagne, qui passerait de 47,5 % à 46 %. Ce bulletin unique permettra le développement d'une politique écologique en matière d'élection. Pour l'élection présidentielle en 2017, 1 300 tonnes de bulletins ont été imprimées, tandis que l'utilisation d'un bulletin unique permettrait de n'en utiliser que 110 tonnes. Cela représente une réduction drastique de la consommation de papier qu'il est important de prendre en considération. Enfin, cette proposition de loi induirait une plus grande égalité entre les partis, en permettant aux petits partis n'ayant pas les moyens d'imprimer eux-mêmes leurs bulletins de figurer sur le bulletin unique. Chacune des cases serait de même taille et l'ordre serait déterminé par un tirage au sort. La

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la propagande électorale est consubstantielle à la pluralité des opinions qui peuvent s'exprimer dans tous les pays démocratiques où le pouvoir n'est pas concentré entre les mains d'un parti unique. Simplifier cette propagande ne doit pas contribuer à museler la diversité et la richesse du débat démocratique. Or le principal fondement de cette proposition de loi, introduit dans l'exposé des motifs, est la multiplication des candidatures aux différents scrutins qui maillent notre démocratie. Après les seize candidats à l'élection présidentielle de 2002, un nouveau record a été établi en 2019, avec pas moins de trente-quatre listes en compétition aux élections européennes. Nous avons tous constaté dans nos communes les problèmes techniques liés à la réception et à la diffusion des professions de foi, des bulletins de vote, mais aussi à la nécessité d'implanter suffisamment de panneaux pour les affiches électorales. D'après les auteurs de cette proposition de loi, le remède consisterait à prendre des mesures adaptatives, voire punitives, potentiellement différentes d'une commune à l'autre, comme l'a expliqué notre collègue Richard. Je dois dire que je ne partage pas, moi non plus, cette vision des choses. Mes chers collègues, interrogeons-nous plutôt sur les raisons de cette forte croissance de pseudo-vocations politiques : personne n'ignore ici que se présenter à une élection nationale confère une visibilité, pour ne pas dire une publicité, que certains saisissent pour satisfaire leur ego à moindres frais. Comme le disait un ancien Président de la République, adepte du mythe socialiste de l'inépuisable source d'argent public, « ça ne coûte rien, c'est l'État qui paie En effet, l'intégralité des frais de campagne est remboursée pour toute candidature recueillant 3 % ou 5 % des suffrages suivant les scrutins, dans la limite de plafonds, mais tellement élevés qu'ils permettent beaucoup d'excentricité. Je pense qu'il conviendrait de revenir sur ces critères, car le financement de tout cela coûte extrêmement cher : entre 26 millions et 89 millions d'euros par élection, comme l'indique un rapport sénatorial de 2015. Je veux bien entendre que la démocratie a un coût, mais nous sommes, dans certains cas, très éloignés de ce noble objectif. Même pour les candidats qui n'atteignent pas le seuil de remboursement, une campagne, c'est-à-dire sans impression de documents électoraux, donne un accès inespéré à des médias nationaux pour diffuser des messages qui ne concernent qu'une partie confidentielle de l'électorat et qui sont même parfois, il faut bien le dire, totalement farfelus. Très sincèrement, je ne crois pas du tout que cela contribue au choix éclairé d'électeurs un peu perdus par une telle dispersion de l'offre. Sans doute faudrait-il tout simplement s'interroger,, sur les conditions qui permettent de se présenter à l'élection européenne ; des filtres ont été comme le nombre et la nature des parrainages. Pour en revenir au texte, une bien curieuse disposition de cette proposition de loi prévoyait des sanctions applicables par les maires à ceux qui ne satisferaient pas à leur déclaration d'affichage au moment de leur déclaration de candidature.

En revanche, implanter le nombre de panneaux correspondant aux déclarations d'intention des candidats d'apposer leurs affiches électorales me semble une idée pertinente, même s'il paraît difficile de prédire la proportion de candidats qui y renonceront effectivement. Une autre disposition m'interpelle particulièrement : la possibilité de réduire la taille des panneaux d'affichage lorsque le nombre de candidatures est supérieur à Nous devons, là aussi, nous interroger sur la faisabilité d'une telle mesure. Cette décision interviendrait à la clôture du dépôt des listes, c'est-à-dire, si on prend l'exemple des prochaines élections municipales, quinze jours avant le premier tour. Cela poserait de sérieux problèmes logistiques à tous les candidats, qui, bien évidemment, auront déjà imprimé leurs affiches. Dès lors, chacun peut imaginer les conséquences pratiques avec des affiches trop grandes pour des formats de panneaux plus petits : un chevauchement bien peu propice à un climat serein entre les concurrents ! Outre ce manque de considération pour le travail de communication des candidats, qui leur demande souvent beaucoup d'énergie, on peut imaginer que cela permettrait en revanche de cacher certaines étiquettes ou soutiens gênants, en quelque sorte « cachez ce soutien que je ne saurais voir » ! Voilà une astuce bien pratique pour masquer des liens qui mettraient à mal les diverses déclarations d'indépendance Pour toutes ces raisons, je proposerai un amendement de suppression de l'alinéa 8 de l'article 1. En définitive, cette proposition de loi aux motivations nobles mais assez fragiles ne me semble pas totalement frappée du sceau du bon sens. le mérite de nous interroger collectivement sur les moyens de faire face à une croissance exponentielle de candidatures aux élections européennes, tout en déplorant par ailleurs la crise des vocations à quelques semaines des élections municipales. Excellent

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons cet après-midi tend à tirer les leçons des élections européennes de mai 2019 pour mieux accompagner les maires dans l'installation des panneaux électoraux et la gestion des bulletins de vote. En effet, pour assurer l'égalité entre les candidats, les communes installent des panneaux électoraux pour l'ensemble des élections, sauf pour les élections sénatoriales, et doivent respecter, à cet égard, des règles très précises concernant la taille, l'ordre et l'emplacement de ces panneaux. Lors des dernières élections européennes, il est apparu qu'un grand nombre de communes ont manqué de panneaux face à la multiplication des candidatures. En effet, trente-quatre listes de candidats se sont présentées, soit treize de plus qu'en 1999. Les panneaux électoraux ne sont pas toujours utilisés par les candidats, alors qu'ils occupent une surface non négligeable de l'espace public. Certains candidats évitent d'imprimer des affiches, notamment parce qu'ils ne pensent pas atteindre le seuil de remboursement de leurs dépenses. listes de candidats aux élections européennes de mai 2019, seule une quinzaine aurait apposé des affiches sur la plupart de leurs panneaux électoraux. C'est pourquoi cette proposition de loi déposée par notre collègue Emmanuel Capus vise à apporter des réponses pratiques à des problèmes constatés au sein de nos territoires. Aussi, pour rationaliser l'utilisation des panneaux électoraux pour l'ensemble des scrutins, l'article 1 de la proposition de loi prévoit deux dispositifs. Le premier vise à faciliter l'organisation du scrutin en renforçant la visibilité des communes. Il s'inspire du droit applicable aux élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants. Désormais, les candidats devraient préciser dans leur déclaration de candidature s'ils souhaitent ou non utiliser des panneaux électoraux. Ces derniers seraient installés à la demande des candidats, et non plus de manière systématique. Le texte prévoit également des sanctions si un candidat réserve des panneaux sans y apposer d'affiches, il devra rembourser à la commune « les frais d'établissement de ces emplacements », dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Le second dispositif tend à optimiser les conditions d'utilisation des panneaux d'affichage. Un décret en Conseil d'État fixerait le nombre et les dimensions des affiches que chaque candidat pourrait apposer sur des panneaux électoraux.

Ainsi, les candidats disposeraient d'un « droit au remords » : ils pourraient solliciter l'installation de panneaux électoraux jusqu'au vendredi précédant le début de la campagne. Cette disposition constitue une souplesse pour les candidats qui modifient leur stratégie électorale en fonction de l'évolution des sondages ou des financements recueillis.

Je suis également satisfait que la commission n'ait pas retenu les mesures visant à réduire de moitié le nombre et la dimension des affiches lorsque les panneaux électoraux sont utilisés par plus de quinze candidats. En effet, cela pouvait conduire à mettre au pilon de nombreuses affiches. S'agissant des élections municipales, seuls quatre jours séparent le dépôt des candidatures et le début de la campagne officielle du premier tour. Beaucoup de candidats sont donc contraints d'imprimer leurs affiches avant de connaître le nombre total de candidatures. Enfin, je me félicite que la commission ait adopté un dispositif plus souple, consacrant la possibilité pour le maire d'adapter les dimensions des panneaux électoraux, à trois conditions premièrement, que le nombre de panneaux à installer soit supérieur à quinze ; deuxièmement, que la commune ne dispose pas d'un nombre suffisant de panneaux ; troisièmement, que tous les candidats bénéficient d'une surface égale pour apposer leurs affiches. Madame la ministre, mes chers collègues, toujours attentif aux préoccupations exprimées par les collectivités territoriales, le groupe Les Indépendants soutient pleinement l'objectif visé au travers de cette proposition de loi. L'ensemble de mon groupe votera donc en faveur de ce texte. La discussion générale est close.

inapplicable sur le terrain, car les délais sont extrêmement courts. Si l'on prend l'exemple des élections municipales- elles vont se dérouler dans quelques semaines -, la date de clôture des déclarations de candidature

Je ne suis pas sûr que l'on se rendre service en rigidifiant de cette façon la législation. Lorsqu'un certain nombre de difficultés apparaîtront, le Gouvernement

la proposition de loi tendait à réduire de moitié la taille de toutes les affiches lorsque les panneaux sont utilisés par plus de quinze candidats. Or cela soulevait des difficultés pratiques, car la plupart des affiches sont imprimées avant le délai limite pour le dépôt des candidatures.

telle faculté serait réservée aux hypothèses où la commune ne dispose pas de suffisamment de panneaux. Elle présenterait le mérite de permettre aux maires de répondre à des problèmes concrets, tout en respectant le droit des candidats.

Cet alinéa ne précise pas dans quelle mesure le maire peut réduire la dimension des panneaux. En l'état du texte, un maire pourrait choisir, en fonction du nombre de candidats, une dimension pour les panneaux qui soit inférieure à la taille des affiches, fixée, elle, par décret. Les candidats pourraient ainsi se retrouver avec des affiches inadaptées aux panneaux mis en place, ce qui porterait atteinte à leur liberté d'expression. En outre, la possibilité laissée au maire de diminuer la dimension des panneaux d'affichage

la rédaction du texte, en prévoyant que les maires ne peuvent restreindre les panneaux quand ils les divisent que dans les limites prévues par voie réglementaire, c'est-à-dire par le fameux décret.

une circulaire pour indiquer aux maires ce qu'ils doivent faire ; de temps en temps, ils aiment bien savoir ce qu'ils ont à faire dans le cadre de ces campagnes qui relèvent de l'autorité du Gouvernement. Puisque nous sommes à peu près tous d'accord, je vous enjoins à voter tous ensemble cet amendement de suppression.

pour réduire la taille des panneaux à leur plus juste proportion, c'est-à-dire au minimum à la taille de l'affiche réglementaire- ni plus ni moins. Il me semble que la commission a fait preuve de sagesse. C'est la raison pour laquelle je soutiens vivement sa version et je

Si j'avais encore quelques doutes, le débat qui vient d'avoir lieu me montre que, moins on en mettra dans ce texte, mieux ce sera

Lors des dernières élections législatives, les candidats de la majorité présidentielle se sont tous affichés sur les panneaux électoraux avec le chef de l'État, dès lors candidat dans les 577 circonscriptions. Or on n'est pas député par procuration. On est élu sur son nom pour représenter les citoyens d'un territoire. Malgré la courte période entre l'élection présidentielle et les élections législatives, la responsabilité politique n'est pas la même. Le Président de la République est le Président de tous les Français, pas le député de tous les Français. L'exécutif ne peut pas se substituer au législatif, ni l'inverse. C'est la sacro-sainte séparation des pouvoirs régulièrement invoquée. Il s'agit insensiblement, mais bien visiblement, d'une dérive de nos principes constitutionnels. Raymond Aron parlait d'« empire parlementaire » pour qualifier la V République. Elle est de plus en plus monarchique, de moins en moins républicaine. Par ailleurs, d'autres candidats choisissent de faire figurer sur leur affiche le leader de leur mouvement. Cette identification à une personnalité nationale, qui n'est pas elle-même éligible sur le territoire concerné, entraîne une forme de confusion, de dépersonnalisation ou, pis, d'anonymisation des candidatures. Afin d'assurer une meilleure lisibilité politique, je propose que ne puissent figurer et être mentionnés sur les affiches et les bulletins de vote que les noms et les photographies des candidats et des suppléants à l'élection visée.

de loi du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral et qui entrera en vigueur le 30 juin prochain.

Heureusement, tout cela a été repris, et bien repris, suivant la vieille tradition de la République. Moi, je voudrais que, selon la vieille tradition de la République, on en revienne à des candidats de terrain, à ceux qui sont réellement élus sur leurs opinions « clairement affichées »- c'est la bonne

élections législatives suivent l'élection du Président de la République. Le Président de la République est devenu le chef de la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Il est donc le chef de tout

dans une démocratie incarnée, que de permettre d'utiliser sa photographie ? Je signale que tous les partis politiques de France ont, tour à tour, utilisé cette faculté après l'élection de leur candidat à la présidence de la République.

Monsieur le rapporteur,

Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. Je rappelle que l'auteur de la demande dispose d'un temps de parole de huit minutes, puis le Gouvernement répond pour une durée équivalente.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à titre liminaire, je souhaite remercier notre collègue Alain Fouché, qui est à l'origine de ce débat. Je me réjouis que notre assemblée se saisisse de cette thématique et mène une réflexion sur la pertinence des outils de régulation du foncier agricole. Dans un ouvrage intitulé, Edgard Pisani écrivait J'ai longtemps cru que le problème foncier était de nature juridique, technique, économique et qu'une bonne dose d'ingéniosité suffirait à le résoudre. J'ai lentement découvert qu'il était le problème politique le plus significatif qui soit parce que nos définitions et nos pratiques foncières fondent tout à la fois notre civilisation et notre système de pouvoir, façonnent nos comportements. La politique foncière agricole s'est construite en France après la Seconde Guerre mondiale afin de permettre à notre pays d'atteindre l'autonomie alimentaire. Elle a permis d'encourager l'investissement et d'accroître la productivité. Elle a été renforcée dès la fin des années 1950 par la création de la PAC. La première véritable politique des structures agricoles est née de la nécessité d'entamer un processus de modernisation de notre agriculture. Elle non seulement sur une politique de marché et de renforcement des filières, mais aussi sur un changement profond des structures d'exploitation agricole. Les lois d'orientation de 1960 et 1962 ont offert un ensemble cohérent de textes visant à infléchir et à encadrer l'évolution des exploitations, changeant ainsi profondément le paysage agricole et rural français.

familiale et établi la parité de revenus entre l'agriculture et les autres activités économiques. Ces transformations supposaient une politique d'aménagement foncier adaptée et des transferts de terres très importants. L'État s'est alors doté d'outils de maîtrise de cette politique foncière. Il s'agissait d'abord de mettre en valeur le droit d'usage au même titre que le droit de propriété. À cette fin, la loi d'orientation de 1960 s'est appuyée sur le statut du fermage, datant de 1946, en le consolidant et en élargissant notamment les possibilités de modernisation de l'exploitation. a encore été complété dans les années 1970, pour conforter la stabilité et la liberté d'investissement des fermiers.

En effet, les enjeux actuels de la régulation foncière sont multiples. Bien entendu, je ne peux que les évoquer rapidement, tout en gardant à l'esprit leur complexité.

Le développement de l'évolution de la structuration en société rend, dans un certain nombre de cas, les outils de régulation du foncier inopérants. On vend et on achète de plus en plus de parts de société, mais de moins en moins de foncier classique. Force est de constater que ce phénomène est encore plus important dans la filière viticole. Les exploitations agricoles sont donc portées, le plus souvent, sous des formes sociétaires, comme les GAEC, les EARL, complétées par d'autres dispositifs sociétaires concernant plus spécifiquement le foncier et l'immobilier, tels que les GFA et les SCI, entre autres structures. Ces évolutions ne sont pas négligeables. D'une part, les Safer et, plus largement, la politique des structures sont limitées quant à leur possibilité d'orientation. transformations ouvrent la voie à une financiarisation croissante du foncier et à des acquisitions extérieures non contrôlées et non régulées. Elles peuvent entraîner des concentrations foncières très importantes, fragilisant ainsi le tissu agricole et viticole. autre phénomène : le mode classique de faire-valoir indirect, qui permet notamment aux propriétaires bailleurs de louer en fermage leurs terres à des fermiers exploitants, est concurrencé par le travail à façon. Les exploitants font ainsi réaliser leurs travaux agricoles par une entreprise. Cette délégation représente aujourd'hui 12 % des exploitations dites « de grandes cultures ». Cela doit nous inviter à réfléchir

au changement climatique et à la gestion de la ressource en eau ; ou encore à d'autres conflits d'usage, en lien avec les énergies renouvelables et les compensations forestières et écologiques, qui sont d'autres sources de pression sur le foncier agricole.

Le notariat français a d'ailleurs consacré son congrès de 2018 au foncier agricole, proposant notamment de fixer de nouveaux objectifs afin d'être en ligne avec les besoins de demain.

Notre politique foncière, depuis près de soixante ans, a permis de bâtir une agriculture moderne performante, diversifiée et présente sur l'ensemble du territoire, avec comme fil conducteur l'autonomie et la souveraineté agricole et alimentaire de notre pays. Mes chers collègues, vous l'avez compris, il y a urgence à se préoccuper de cette question. C'est la raison pour laquelle les élus du groupe Les Indépendants ont souhaité l'inscrire à l'ordre du jour du Sénat. Faisons le voeu que ce débat nous permette d'abord d'évaluer la pertinence des outils de régulation et, ensuite, de trouver les solutions pour les améliorer et les adapter aux réalités d'aujourd'hui. Il faut limiter les excès tout en laissant à la liberté d'entreprendre toute sa place et sa créativité. Très bien ! C'est aussi l'une des qualités de la France et de son expression dans le monde. Ainsi, une ligne de crête est à trouver, et notre système doit Mais comme le disait Edgard Pisani : « Cessons de toujours mettre en avant les difficultés à faire les choses et prenons plutôt en compte, avant tout, la nécessité de les faire !

en vue d'assurer la stabilité des structures foncières des exploitations agricoles en location et de garantir au fermier le bénéfice de ses gains de productivité par la limitation des loyers. le statut du fermage a garanti l'équilibre des relations bailleurs-preneurs. Dans les années 1960, l'instauration du contrôle des structures et la création des Safer ont répondu aux enjeux de renouvellement des générations et de consolidation d'exploitations viables dans les territoires.

Cette consultation était un préalable indispensable, car, j'insiste sur ce choix de méthode, il est hors de question que seuls les parlementaires travaillent sur ces outils ; la profession agricole doit être le plus largement, le plus unanimement possible

la parole est à Mme Noëlle Rauscent. Chacun sait que l'accès au foncier reste difficile pour les agriculteurs qui souhaitent s'installer : les fermes sont de plus en plus grandes et les terres agricoles, qui représentent une valeur refuge pour les financiers, sont de plus en plus convoitées.

qui menace notre souveraineté alimentaire. Dans ce contexte, toute nouvelle décision de passer d'une terre agricole à une zone constructible doit être justifiée par une réelle nécessité. De plus, nous devons freiner le développement des panneaux photovoltaïques au sol et favoriser leur installation sur les bâtiments agricoles. Par ailleurs, nous observons un réel besoin de moderniser le contrôle des structures. Les départements, qui sont au plus près de nos territoires, sortent perdants des nouveaux schémas de régulation. Comme j'ai pu l'entendre, les CDOA ne sont plus que des chambres d'enregistrement

Mais le contrôle des structures et le statut du fermage sont fragilisés par la progression de montages sociétaires destinés à échapper au contrôle, l'accaparement du foncier par des investisseurs étrangers, l'installation d'activités de loisir et de nouvelles formes d'exploitation conduisant à l'éviction des agriculteurs. La profession ne milite pas pour une refonte complète de ces outils, mais pour leur rénovation mesurée et leur renforcement. Seule une définition de l'agriculteur actif professionnel,

était un moyen de reconnaître à sa juste valeur le labeur des agriculteurs, pourquoi pas ? Si cette nouvelle définition permettait à ceux qui labourent la terre d'être revalorisés, pourquoi pas ?

Pour remédier à la disette alimentaire consécutive à la Seconde Guerre mondiale, un grand programme de modernisation de l'agriculture française a réaménagé le territoire agricole au service d'une agriculture pétrolière utilisant sans limites les matières et les énergies fossiles. 20 000 remembrements ont été financés, 500 000 kilomètres de haies supprimés, des milliers de champs drainés ou irrigués, des milliers de mares supprimées, des centaines de kilomètres de cours d'eau rectifiés et des milliers d'hectares de zones humides retournés. Les sols ont été massivement artificialisés et continuent de l'être à un rythme soutenu. La taille des parcelles s'est accrue. Les rendements ont certes augmenté grâce aux engrais et aux pesticides, mais on mesure aujourd'hui la contribution de ceux-ci aux pollutions de toute sorte et, bien sûr, au réchauffement de la planète. La note, assurément, sera Aucun insecticide n'est aussi efficace que l'oiseau, la coccinelle ou la grenouille qui loge dans les arbres, les fossés, les mares, les prairies humides que, malheureusement, l'intensification agricole de l'ère du pétrole a rasés, comblés, retournés ou abandonnés. Il ne faut pourtant pas désespérer : dame nature est bonne fille ... Le projet d'industrialisation de l'agriculture comportait le volet essentiel de l'aménagement foncier. Aujourd'hui, l'heureuse réorientation de l'agroécologie appelle un nouveau projet spatial, qui en accompagne et favorise la mise en oeuvre. Une loi foncière est attendue. À cet égard, j'ai bien entendu le questionnement pertinent de mon collègue et ami Franck Menonville.

Dans le cadre de la réforme de la PAC, la création et l'entretien de ces structures paysagères et écologiques pertinentes devraient faire l'objet de paiements pour services environnementaux dans tous les bassins de notre pays, avec le concours des agences de l'eau. Qu'en pensez-vous ? La parole est à

au glyphosate, une autre molécule permettant à l'agriculture de conservation de continuer à se développer, il faudrait continuer avec le glyphosate.

monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement n'est pas resté sans agir, notamment en vue de détecter le plus en amont possible de telles acquisitions par des personnes, physiques ou morales, non ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne.

aujourd'hui aux outils de régulation du foncier de ne pas avoir empêché l'artificialisation des surfaces agricoles et de ne pas permettre le renouvellement des générations, ainsi que l'essor de nouvelles modalités d'exploitation prenant en compte les enjeux environnementaux liés à l'activité agricole.

à celle de nombreux élus, le devenir des 670 hectares du triangle de Gonesse, dernière niche agricole aux portes de Paris, reste soumis à des menaces de bétonisation. un autre quartier d'affaires ? Ou, comme l'a annoncé Emmanuel Macron, plusieurs projets coordonnés sur une superficie plus étendue, plus mixte et plus moderne se pose également de l'évolution du type de cultures sur ces 670 hectares aujourd'hui cultivés par une dizaine d'exploitants, qui ne sont pas tous propriétaires des terres. Blé, colza, orge, maïs : autant de productions qui ne sont pas forcément en rapport avec la consommation du territoire qui entoure cette poche agricole. Or, comme il a été rappelé lors des débats publics et réunions sur la préservation et l'avenir de ces terres agricoles, il n'y a pas si longtemps que la culture maraîchère et fruitière prédominait encore, assurant l'autosuffisance des villes alentours. Certains projets visent à y revenir pour développer une agriculture au service des agriculteurs, des consommateurs et de l'environnement, par la promotion des circuits courts au plus près du lieu de production ; je pense, par

la ressource de ce sol est absolument indispensable. La position du Gouvernement est très claire : non au grand projet EuropaCity ; nous verrons s'il y a d'autres projets,

Pourtant, ce sujet est au coeur de la place et des moyens que la société française doit donner à son agriculture et à l'exercice de la profession d'agriculteur. Parmi les multiples enjeux posés, en voici quelques-uns qui permettent de mesurer l'importance et l'urgence de la protection et la valorisation du foncier agricole, la diversité des formes d'exercice de la profession d'agriculteur, la contribution des agricultures à la biodiversité et à la préservation de l'environnement,

de présenter un projet de loi de régulation du foncier agricole, dont les principes ne reposeraient plus sur des critères techniques, comme c'est le cas aujourd'hui, mais sur les objectifs des politiques publiques qui touchent à l'emploi et à l'installation des jeunes, aux attentes des consommateurs et des élus locaux, à la transition agroécologique, à la biodiversité et au développement des territoires

de contrôle sur toutes les cessions de parts de sociétés, hors opérations intrafamiliales, et un pouvoir de négociation dans les cas problématiques au regard des enjeux de concentration et de respect des politiques territoriales ? La parole est à M. le ministre.

La maîtrise du foncier agricole relève de la souveraineté nationale. Les Safer doivent être au coeur de cette régulation publique modernisée. Leur relation avec le contrôle des structures doit être revue, la mutation de parts sociales devant donner lieu à un agrément répondant aux objectifs d'un cahier des charges. Enfin, une évaluation des résultats de cette régulation modernisée doit être périodiquement réalisée.

du foncier agricole. Ils représentent une spécificité nationale, dont la France peut être fière. J'appelle donc depuis des mois l'attention sur les problèmes de budget rencontrés par certaines Safer et les difficultés qui en découlent dans la mise en oeuvre de leurs missions de service public. Cela les a déjà conduites à déstocker le foncier qu'elles avaient en réserve, et la situation ne cesse de se détériorer dans un contexte de hausse des prix du foncier. Les Safer jouent un rôle essentiel dans l'aménagement du territoire et la politique agricole nationale. En parallèle, les établissements publics fonciers régionaux poursuivent une mission de maîtrise foncière. Lorsque leurs réserves foncières sont agricoles, les missions de la Safer et des EPF se recoupent. Il existe déjà un terrain d'entente et de coordination sur certains territoires.

Les Safer intervenant dans la partie agricole des missions des EPF, un transfert de ressources pourrait s'avérer pertinent. Enfin, je tiens à rappeler que les Safer font face à un manque d'information important concernant les ventes de biens fonciers, ce qui ne peut que nuire à leur activité.

Elle permet notamment un partage de la valeur ajoutée entre les acteurs répartis sur les territoires grâce à un maillage de petites exploitations. La fiscalité patrimoniale, que ce soit celle sur les successions ou celle sur les donations, frappe lourdement les transmissions familiales, notamment lorsque le prix du foncier est élevé. En conséquence, les héritiers sont incités à céder ce foncier, plutôt qu'à le conserver ou à le louer à des membres de la famille, ce qui fait courir un risque de morcellement et de disparition des exploitations familiales. Par exemple, entre 2006 et 2016, une diminution de 6 % des structures moyennes a été constatée en Champagne. Les mesures actuelles, principalement l'exonération partielle des biens loués par bail à long terme, n'apparaissent plus suffisantes pour résoudre ce problème. Monsieur le ministre, j'aimerais recueillir votre avis sur quelques propositions- j'ai porté certaines d'entre elles lors de l'examen du premièrement, favoriser les transmissions dans un cadre familial au travers d'une exonération significative des droits de donation et de succession pour les biens loués pendant une durée longue exonérer d'impôt sur la fortune immobilière les propriétaires qui affectent durablement leurs terres à des exploitations agricoles ; troisièmement, rendre le contrôle du foncier plus efficient, lorsque sa mutation prend la forme d'une vente de droits démembrés ou d'une cession de parts de société ; quatrièmement, rétablir une fiscalité patrimoniale incitative pour les investissements dans les parts de groupements fonciers agricoles. La parole

premièrement, triplement du plafond d'exonération des droits de succession ou de donation lors de la transmission de biens loués par bail à long terme ; deuxièmement, élargissement du crédit vendeur, qui permet d'étaler l'imposition des plus-values lors des cessions.

même rappeler le rapport de la Cour des comptes de 2014, qui pointait des dérives, notamment un dévoiement de leurs missions traditionnelles au profit de pratiques communément appelées opérations de substitution. Il s'agit d'opérations qui n'ont strictement rien à voir avec les missions initiales des Safer, à savoir le remembrement et l'installation des jeunes et qui permettent aux acquéreurs de ne pas s'acquitter des droits fiscaux, dont les Safer sont exemptées, et à ces dernières de toucher une commission en échange. échange. Selon la Cour des comptes, le coût fiscal de ces opérations s'élève à plus de 45 millions d'euros, les perdants étant les départements et les communes ... La Cour constate par ailleurs que cet avantage fiscal concerne de plus en plus d'opérations relatives à des biens ruraux bâtis qui n'ont strictement rien à voir avec les biens agricoles. Je vous invite, monsieur le ministre- j'en ai encore fait l'expérience tout à l'heure à aller sur le site internet géré par la Fédération nationale des Safer ; vous y trouverez des résidences secondaires qui n'ont aucune terre agricole autour.

je ne suis pas certain que la combinaison du droit de préemption, de la politique des structures et des mécanismes de fixation des loyers soit un véritable élément d'attractivité. Qu'envisagez-vous de faire pour que les investisseurs n'hésitent pas à investir en milieu rural ?

L'objectif des SCOT, des PLUI ou des PLU est clairement d'optimiser la consommation des espaces, en préservant au mieux le foncier agricole et viticole. Ainsi, en Gironde, le concept de trame pourpre, à l'instar des trames bleues et vertes, permet, sans en avoir la même force, d'améliorer la prise en compte des enjeux viticoles pour la rédaction des documents d'urbanisme, mais nous sommes clairement confrontés à une incapacité d'agir pour combler les dents creuses viticoles en milieu urbain ou en périphérie. Cet objectif louable permettant notamment de rationaliser les périmètres et les bandes de protection ne dispose pas d'outil opérationnel de négociation et de compensation. Il est en effet légitime que, dans cette perspective, toute consommation foncière viticole, notamment en appellation d'origine contrôlée, soit compensée pour maintenir les surfaces d'exploitation, mais ces outils de compensation sont aujourd'hui quasi inexistants ou inopérants. Il serait judicieux d'établir sur ces sujets des coopérations fonctionnelles entre les Safer et les établissements publics fonciers pour créer les moyens de la négociation et de la compensation, que celle-ci soit en nature ou financière. Cet outil de médiation est aujourd'hui essentiel pour optimiser les démarches d'urbanisme, en respectant toutes les parties prenantes. Il serait essentiel pour répondre aux enjeux environnementaux et faciliter l'acceptabilité des projets. Face à l'impuissance actuelle, quelles propositions d'outils de compensation et de médiation foncière pourriez-vous faire pour résoudre nombre de conflits et tensions liés aux proximités viticoles et urbaines ?

Il devient donc urgent de créer des instruments de médiation pour faciliter leur conception et leur approbation, en respectant l'ensemble des parties prenantes. La parole est à M. Cyril Pellevat.

Il faut d'emblée souligner l'importance de la politique foncière en France. Elle représente un atout pour la compétitivité et la durabilité de notre agriculture. À ce titre, cette politique publique mérite d'être préservée et consolidée.

doit être amélioré pour mieux préserver nos terres face à l'accaparement par des investisseurs étrangers. L'un de nos objectifs communs, mes chers collègues, étant de permettre aux agriculteurs d'acquérir progressivement les terres qu'ils exploitent, de ce point de vue où en est le dispositif Sapin, qui vise à mieux appréhender l'acquisition par des pays étrangers des terres agricoles françaises. Je crois qu'il nous faut préserver, renforcer et moderniser les outils de régulation de notre politique foncière agricole. Je terminerai par le cas précis du mitage des terres.

Ce livret vert pourrait être créé sur le modèle du livret A ou du livret de développement durable. Cette idée est portée depuis le début des années 2010 sur différents bancs de l'Assemblée nationale et différentes travées du Sénat. Récemment, dans leur rapport de la mission d'information sur le foncier agricole rendu en décembre 2018 à l'Assemblée nationale, Anne-Laurence Petel et Dominique Potier en ont fait l'une de leurs propositions, mais nous pouvons aussi nous rappeler qu'en 2015 une proposition de loi déposée par une partie de nos collègues du groupe Les Républicains reprenait également le principe de ce livret vert. Ce livret vert présenterait selon moi un triple avantage. Le premier serait de renforcer la lutte contre la pression foncière et l'artificialisation ou l'accaparement des terres agricoles. Il pourrait financer une politique de prêts bonifiés fléchés visant à favoriser l'accès au foncier agricole pour encourager l'installation et le renouvellement des générations. Il pourrait bénéficier aux agriculteurs, mais aussi aux collectifs citoyens et aux collectivités territoriales. Le deuxième avantage, c'est qu'il répondrait à une attente sociétale de plus en plus forte des Français de s'engager vers des politiques plus respectueuses de l'environnement et une alimentation plus sûre. Le troisième avantage que j'identifie viendrait également répondre à une attente forte des Français : avoir accès à une épargne sûre. Monsieur le ministre, la loi sur le foncier agricole tardant à venir et la création de ce livret vert relevant davantage d'une loi de finances, pouvez-vous nous indiquer si le Gouvernement est prêt dans le cadre du prochain projet de budget à accepter le principe de la création de ce livret vert ?

Elle représente en moyenne 27 000 hectares par an, soit l'équivalent de trois à cinq stades de football par heure. De plus, si elle a été divisée par deux entre 2007 et 2017, elle est repartie à la hausse depuis 2015. Dans un rapport publié l'été dernier, France Stratégie estimait pour sa part qu'atteindre l'objectif de « zéro artificialisation nette » dès 2030 nécessiterait de réduire de 70 % l'artificialisation brute et de retourner à la nature 5 500 hectares de terres. L'agriculture est souvent doublement touchée, par l'emprise des ouvrages construits puis par la mobilisation du foncier pour la mise en oeuvre des mesures de compensation environnementale. La reconquête des sols et des friches urbaines peine à se mettre en place, notamment parce qu'elle est coûteuse. L'application de la séquence « éviter-réduire-compenser », présentée comme la solution pour concilier aménagement et environnement, ne semble pas non plus donner les résultats escomptés. Le rôle des Safer comme régulateurs de la consommation du foncier agricole apparaît également de moins en moins prégnant. Aussi, en quoi la loi foncière en préparation sera-t-elle de nature à apporter des solutions à la hauteur de cette consommation inexorable du foncier agricole, notamment en matière de réhabilitation des friches urbaines ?

Nous constatons aussi que certaines fermes laitières sont reprises pour y étendre ou y installer des haras de chevaux de courses appartenant à des sociétés financières françaises ou étrangères. Dans ces deux cas, la terre peut être vendue jusqu'à 20 000 euros l'hectare. Avec un chiffre d'affaires de 1 300 euros par hectare et un bénéfice de l'ordre de 450 euros par hectare, il est impossible pour un jeune agriculteur d'acquérir ces terres et de vivre décemment de son travail. Pourtant, à l'échelle du pays, il est primordial de conserver une indépendance agricole et de produire suffisamment pour nourrir la population : cela a été suffisamment répété au fil de cette journée. L'installation des jeunes agriculteurs doit donc être suivie et encouragée.

Les Safer font aussi l'objet de nombreuses critiques quant à la préemption et à l'attribution des terres, mais aussi quant à leur financement, depuis le retrait du soutien de l'État en 2017. Monsieur le ministre,

le défi du renouvellement des générations et du remplacement des agriculteurs partant à la retraite. Dans ce contexte, la politique de régulation de l'exploitation du foncier le contrôle des structures apparaissent secondaires. N'est-il pas plutôt nécessaire de trouver des agriculteurs, autrement dit de susciter des vocations, plutôt que de s'arc-bouter sur l'attribution la plus égalitaire possible du droit d'exploiter le foncier entre les agriculteurs en place, alors même qu'une exploitation agricole repose sur un projet économique permettant de dégager un revenu décent, et non sur un nombre d'hectares de ce nouveau contexte foncier et de ces enjeux, ne croyez-vous pas nécessaire, monsieur le ministre, de simplifier les conditions d'application du contrôle des structures, dès lors que, dans la plupart des régions, il n'y aura pas pénurie de terres à cultiver et que la réussite d'une entreprise agricole dépend peu de son nombre d'hectares ? Jugez-vous nécessaire de faire des installations, tout particulièrement celles de jeunes non issus du milieu agricole, une priorité, dès lors qu'elles sont indispensables au renouvellement des générations d'agriculteurs ? ? Enfin, estimez-vous possible de mieux maîtriser les agrandissements excessifs en contrôlant plus efficacement les prises de participation dans les sociétés d'exploitation ?

dans le cadre de la concertation, de simplifier le contrôle des structures pour le concentrer sur les opérateurs à enjeu. Ce contrôle est évidemment indispensable, mais nous voulons le faire évoluer. Enfin, concernant là encore l'installation des jeunes,

Avec lui, les physiocrates fondaient leur réflexion économique et politique sur la valorisation du foncier agricole, terreau fertile pour nos libertés individuelles. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui se trouvait donc déjà au fondement de notre développement économique, et sur ce fondement s'enracinaient deux piliers qui structurent encore notre société : la propriété privée des moyens de production et la liberté d'entreprendre. La question du foncier agricole, si elle demeure d'une actualité décisive pour nos agriculteurs, se trouve cependant aujourd'hui en tension avec les grands enjeux de notre siècle, au premier rang desquels figure bien évidemment le défi climatique. Cette question intéresse donc bien au-delà du monde agricole. Elle fait surgir des problèmes nouveaux qui appellent de solutions nouvelles. Et pour cause : les termes du débat ont radicalement changé depuis la fin du XVIII siècle. Comme cela a été rappelé au cours du débat, la question du foncier agricole doit trouver à s'articuler avec notre capacité collective à nous alimenter, à opérer la transition énergétique, à préserver les écosystèmes, à fournir des logements pour une population en croissance continue, à recevoir des infrastructures pour le développement des nouvelles technologies, à faciliter la mobilité de nos concitoyens et, bien sûr, à garantir des revenus décents pour nos agriculteurs. Cet inventaire à la Prévert ne peut que renforcer une conviction que- j'ose le croire -nous partageons tous sur ces travées : la question du foncier agricole est d'une complexité rare. Elle fait se conjuguer, parfois de manière conflictuelle, des objectifs que nous aimerions pouvoir poursuivre de manière parallèle. Cette complexité nous oblige ainsi à opérer des choix difficiles. C'est pour cette raison que notre groupe a opté pour un débat plutôt que pour une proposition de loi. Non qu'un texte de loi ne soit pas nécessaire pour répondre aux défis que nous avons collectivement identifiés- je crois en effet qu'une action législative sera tôt ou tard indispensable plutôt que la question du foncier agricole est trop complexe pour que l'on puisse prétendre la résoudre par des solutions trop simples. Notre travail parlementaire a déjà permis d'identifier de nombreuses pistes d'action pour préserver et valoriser le foncier agricole. Le Gouvernement a également précisé sa vision des problèmes sous-jacents et les solutions qu'il entend mettre en oeuvre. Enfin, les acteurs de terrain se mobilisent dans les territoires pour nous faire remonter leurs opinions et leurs propositions sur la question. Afin de préserver nos terres agricoles et de limiter l'artificialisation de nos sols, le législateur devra très certainement veiller à ce que la Nation protège ce foncier au même titre qu'elle s'attache déjà à protéger la biodiversité et les forêts de notre pays, en refusant de hiérarchiser ces priorités. Telle est l'ampleur de la tâche qui se trouve devant nous. Nous devrons nous y atteler rapidement. Mise en valeur du foncier agricole, portage, transmission, rénovation de la régulation, retraites anticipées, fluidification du dialogue entre les différentes parties prenantes du terrain : les sujets ne manquent pas et ils intéressent le Sénat au premier chef. Le groupe Les Indépendants poursuivra ses travaux dans ce sens afin d'apporter des solutions concrètes aux défis du foncier agricole. Pour l'heure, je voudrais remercier chaleureusement nos collègues de tous les groupes pour leur participation à ce débat. Je voudrais vous remercier plus particulièrement, monsieur le ministre, pour les réponses que vous nous avez apportées sur les sujets que j'évoquais à l'instant et sur bien d'autres. Je voudrais enfin remercier nos collègues Alain Fouché et Franck Menonville, à l'origine de ce débat dont nous voyons bien, à son issue, à quel point il était nécessaire. Nous en